une heures : Suite du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification

En 2014 comme en 2020, les maires et les présidents d'intercommunalité ont fait obstacle à ces transferts, non pas au motif que leur objectif n'était pas souhaitable, mais parce que le cadre juridique compliquait l'effectivité des décisions prises par les présidents auxquels étaient transférés des pouvoirs de police. Sans modifier le code de l'environnement, le présent amendement vise à permettre au président de l'intercommunalité, en complément des possibilités d'ores et déjà prévues par ce code, de missionner d'autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de gestion des déchets sauvages. La parole

Cet amendement, déposé par notre collègue Ronan Dantec, vise à élargir la liste des agents pouvant être assermentés en matière de police des déchets. Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires au président de l'intercommunalité vise à favoriser la cohérence entre l'exercice par cette dernière de ses compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer. À de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et les présidents d'intercommunalité ont fait obstacle à ces transferts, non pas au motif que leur objectif n'était pas souhaitable, mais parce que le cadre juridique compliquait l'effectivité des décisions prises par les présidents auxquels étaient transférés des pouvoirs de police. Cela est particulièrement marqué pour les attributions correspondant aux domaines de la collecte des déchets et de la gestion des déchets sauvages. En effet, le code de l'environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions en la matière sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales- agents des douanes ou de la répression des fraudes -ou ne le sont que par celles qui disposent d'importants moyens- agents de police judiciaire adjoints ou encore médecins territoriaux. Sans modifier le code de l'environnement, le présent amendement permettre au président de l'intercommunalité, en complément des possibilités d'ores et déjà prévues par ce code, de missionner d'autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de gestion des déchets sauvages.

corrige la rédaction de l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement pour permettre au président d'un groupement de collectivités territoriales

Le dispositif s'articulerait de la manière suivante : sur son territoire, la métropole participerait à l'élaboration du programme opérationnel régional. Dans l'hypothèse où un accord n'est pas trouvé avec la région, les orientations de les décisions sont alors prises en tenant compte du programme régional. La métropole déterminerait notamment son propre dispositif de stratégie territoriale intégrée. Pour que les décisions qui découlent de ces programmes régionaux soient opérationnelles, il est nécessaire qu'un véritable dialogue entre les régions et les métropoles soit instauré. Plus que jamais, il faut affirmer le caractère indispensable du partenariat entre métropoles et régions dans la mise en place de ce dispositif spécifique de coélaboration et de coadoption des programmes opérationnels régionaux. Quel

Toutefois, le dispositif proposé reviendrait à subordonner à l'accord de la métropole les choix faits par la région pour la gestion des fonds européens

à l'élaboration du plan de mobilité les autorités organisatrices équivalentes des pays voisins. L'article 58, tel qu'il figurait dans permettait d'intégrer la question des transports de personnes et de marchandises dans les échanges transfrontaliers. Le plan de mobilité détermine les principes qui régissent l'organisation de la mobilité des personnes et des marchandises, de de la circulation et du stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice. Il est actuellement élaboré en tenant compte de la diversité des composantes des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités limitrophes. Dans les territoires frontaliers, nous souhaitons que soit formalisée la possibilité d'associer à cette élaboration les autorités organisatrices équivalentes des pays voisins, une fois celles-ci identifiées. Quel

rectifié . L'élaboration des Sraddet constitue un processus lourd et complexe, qui mobilise du temps et un budget important pour les régions. Dans la perspective des changements introduits par le projet de loi Climat et résilience, ces schémas devront en outre être prochainement révisés pour intégrer diverses obligations.

il apparaît opportun d'assouplir le cadre actuel en remplaçant l'enquête publique imposée pour cette révision par une consultation du public, dont les modalités seraient fixées par le conseil régional. Tel est l'objet du présent amendement.

de les y autoriser par la loi. Les collectivités étrangères peuvent donc parfaitement être consultées par une commune, voire une intercommunalité, sur le projet de PLU. En revanche, ces amendements tendent également à accorder à ces collectivités étrangères le droit d'être consultées si elles le demandent, ce qui ne me paraît pas opportun.

la partie réglementaire du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de consulter les collectivités territoriales des États limitrophes ou tout organisme étranger compétent en matière d'aménagement, d'environnement ou encore d'architecture. La disposition que vous proposez

une meilleure cohérence entre eux. Rappelons quelques éléments de contexte. Partout dans le monde, les études convergent pour souligner l'importance fondamentale du facteur environnemental dans les décès prématurés et l'émergence de maladies. Une étude de l'université Harvard parue en 2021 établit que 8 millions de personnes sont mortes prématurément en 2018 à cause de la pollution de l'air. Au total, l'OMS estime que près de 14 millions de décès sont liés chaque année à des facteurs environnementaux tels que la pollution de l'air, de l'eau ou des sols, ou encore l'exposition à des substances chimiques, qui provoque une centaine de maladies chez les humains. Cela représente 24 % des décès dans le monde, soit près La France n'est pas épargnée. Selon l'OMS, 14 % de la mortalité annuelle prématurée dans notre pays est due à des causes environnementales. Cela représente environ 84 000 morts

H5N1, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 -dues à la dégradation de l'environnement et à la perte de la biodiversité transforment la santé environnementale en un sujet majeur pour les pouvoirs publics et les collectivités. C'est dans ce contexte que nous proposons de renforcer le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en précisant ses liens avec le plan régional santé-environnement et en inscrivant dans la loi qu'il devra être compatible avec les objectifs et les mesures prévus par ce plan. Ce que nous cherchons Ce que nous cherchons à garantir par cet amendement, c'est la cohérence des politiques locales de santé, une cohérence désormais requise pour l'efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre les effets du dérèglement climatique sur la santé, qui est un enjeu majeur du XXI siècle. Quel

au contraire, cela permet de définir de manière plus claire un certain nombre d'objectifs communs et de lignes d'horizon vers lesquelles il faut tendre. La parole est à Mme la ministre.

territoriales de manière à rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l'élaboration des Sraddet, cette consultation étant aujourd'hui

n° 304 rectifié, nous demandons la suppression pure et simple de l'article 59, qui pose un sérieux problème d'indépendance et de continuité. La version adoptée par notre commission des lois ne fait que renforcer le caractère problématique de cet article suscite des interrogations majeures. En effet, près d'un tiers des citoyens de l'Union européenne vivent ou travaillent dans des régions frontalières. En France, 355 000 de nos concitoyennes et concitoyens traversent la frontière pour aller travailler ; ils sont dix fois moins à faire le chemin dans le sens inverse. Ces mouvements de population engendrent notamment la nécessité de renforcer nos infrastructures infrastructures de transport. Votre réponse aux pertes de revenus et aux nécessités d'investissement dans les infrastructures et dans d'autres services publics serait d'étendre le financement étranger de ceux-ci. Cela nous Sur toutes les travées, j'entends la préoccupation de permettre aux collectivités, notamment locales, d'être au coeur de la relance de l'économie. Les SPL sont une des personnes morales qui doit participer à cet effort, partout en France. Néanmoins, la captation par des entreprises étrangères de l'argent public pour réaliser des missions d'intérêt général qui relèvent de nos collectivités locales n'est pas acceptable. On comprend bien l'intérêt de cette situation : partager la note pour les projets d'aménagement. Ce type de raisonnement risque bien d'engendrer une diminution du bénéfice de la commande publique pour les entreprises de notre pays,

L'argument est encore plus flagrant dans le cas d'une prise de contrôle étrangère d'une SPL. Outre l'argument de l'activité économique et de l'emploi, qu'adviendra-t-il du service public le jour où l'actionnariat étranger disparaîtra ? Il n'y a là aucune garantie. L'étude d'impact est très claire à cet égard : « La cessation d'activité de la société peut peut conduire à l'interruption d'un service public concédé ou d'une opération réalisée sous mandat. Dans ce cas, la collectivité peut être placée en situation de reprendre elle-même le service public ou l'opération inachevée, générant ainsi d'importantes charges financières. »

Le texte de la commission a supprimé la limitation des capitaux des collectivités étrangères dans les sociétés publiques locales transfrontalières, afin de faciliter la constitution de sociétés rassemblant des collectivités de trois nationalités différentes. La règle instaurée par le Gouvernement, qui est d'ailleurs celle qui s'applique depuis des années aux SEML transfrontalières, vise à protéger les collectivités territoriales et groupements français qui constitueraient de telles sociétés. En effet, les SPL sont des sociétés anonymes, dont la détention du capital confère un nombre proportionnel de voix dans la société, lequel nombre détermine la capacité à décider. Permettre que la participation des collectivités territoriales françaises puisse être réduite à une simple minorité de blocage, dans le meilleur des cas, les expose au risque de se voir imposer des décisions auxquelles elles s'opposent. La majorité du capital et des voix dans les organes délibérants des sociétés est la garantie que nos collectivités ne pourront pas se voir imposer des décisions qu'elles jugeraient contraires à la bonne gestion de leur service public et à l'intérêt public local. De plus, aucun projet nécessitant la constitution d'une SPL tripartite n'a été signalé. Enfin, l'objet social de ces SPL a été étendu. Si la logique de cette extension peut se comprendre, elle ne doit pas permettre la constitution de SPL transfrontalières dont l'objet social inclurait une ou plusieurs activités ne relevant de la compétence

La commission a estimé ce plafonnement inutilement rigide. Il pourrait bloquer, par exemple, la constitution de SPL associant des collectivités de trois pays. L'argument du Gouvernement selon lequel notre rédaction permettrait à des collectivités françaises de se voir imposer des décisions contre leur gré ne tient pas. Tout d'abord, les collectivités françaises sont d'ores et déjà autorisées par la loi à participer au capital de sociétés étrangères, au sein desquelles rien ne garantit aient le dernier mot. Ensuite, si tous les États raisonnaient ainsi, la constitution de SPL associant des collectivités de plusieurs pays deviendrait tout simplement impossible. Enfin, il appartient aux collectivités associées de déterminer librement, dans les statuts de la société, les modalités de prise de décision adéquates. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable

du bon sens ... Selon nous, cet amendement, qui vise à subordonner les prises de participation de collectivités locales étrangères au capital d'une SPL

à que les collectivités territoriales ne puissent avoir de coopération qu'avec les États qui entretiennent des relations diplomatiques avec la France. Cela ne me semble pas constituer une disposition très lourde ni très compliquée.

Si on peut considérer l'objectif comme légitime, il semble que la rédaction proposée ne l'atteigne pas. La France entretient, par exemple, des relations diplomatiques avec la Russie, bien qu'elle ne reconnaisse pas la souveraineté de cette dernière sur la Crimée ni, par conséquent, les autorités actuelles de Crimée. À vrai dire, je pense que l'amendement est satisfait par le droit en vigueur, car, lorsque la loi parle d'« autorités locales étrangères », elle désigne nécessairement des autorités locales reconnues légitimes par le gouvernement français, seule autorité de la République habilitée à procéder à des actes de reconnaissance internationale.

territoriales, l'action internationale des collectivités territoriales et de leurs groupements est soumise au « respect des engagements internationaux de la France ». Ainsi, il n'est pas possible, pour des collectivités ou leurs groupements, d'entretenir des relations avec une autorité locale étrangère

départemental de coopération transfrontalière que seraient désormais chargés d'élaborer tous les départements frontaliers. Cela ne semble pas, selon nous, faire sens, car ce schéma constitue la traduction opérationnelle du chef de filât reconnu aux départements concernés en la matière. Or je rappelle que la responsabilité de chef de file, définie par le CGCT, ne concerne que la coopération entre collectivités territoriales et non entre ces dernières et l'État ou d'autres personnes chargées de missions de service public. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

l'ajout suivant : « ainsi que l'organisme de liaison mentionné à l'article [ ...] du code de la sécurité sociale en lien avec les organismes nationaux de sécurité sociale et son homologue du pays concerné.

C'est dans cette perspective que cet article accélère et renforce le partage d'informations entre les services de l'administration, et ce par une simplification de la mise en oeuvre du dispositif « dites-le-nous une fois sous le contrôle rigoureux de la CNIL, avec laquelle nous avons eu des échanges fructueux. Le partage de données entre l'État et les collectivités existe déjà dans le cadre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration 280 collectivités sont déjà raccordées aux données du quotient familial de la CAF et du revenu fiscal de référence de la DGFiP pour simplifier les demandes d'inscription à la cantine ou à la crèche en calculant les remises tarifaires 803 collectivités utilisent FranceConnect pour simplifier la connexion de leurs administrés. Toutefois, les règles actuelles prévoient un système où les échanges ne sont autorisés que dans des cas précis et pour des données précises décidés au niveau réglementaire. L'idée initiale de l'article était d'inverser le paradigme en faisant du partage de données entre administrations la règle par défaut, plutôt que l'exception, en supprimant la liste limitative de données et procédures pouvant faire l'objet d'un partage, tout en désignant des administrations de référence pour chaque type de données.

à la version initiale de l'article.

divers organismes publics. Certes, elles font partie de l'administration publique territoriale. Il n'en demeure pas moins que les plus petites de nos collectivités font aussi face à des difficultés concrètes et pratiques, similaires à celles de nos administrés.

centralise, sur un seul site internet, toutes les aides pour accompagner les projets des collectivités territoriales.

au bénéfice de l'usager. La complexité administrative éloigne du service public ceux qui en ont le plus besoin. Une des complexités principales rencontrées par les usagers est de devoir fournir, lors de leur demande, des données ou informations déjà détenues par les administrations leur revenu fiscal de référence, leur quotient familial, leur justificatif de certificat d'immatriculation, etc. L'objectif de cette mesure est de faire en sorte que les administrations s'échangent les informations, au lieu de les demander à l'usager lors de leur démarche.

ou de manière proactive, toujours dans le seul intérêt de l'usager, et en lui permettant de s'opposer à la poursuite du traitement à chaque fois. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un partage de données dans une autre finalité. La mise en oeuvre de ce dispositif d'échange de données pour cette nouvelle finalité est strictement encadrée par le présent article. Par ailleurs, l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration prévoit déjà qu'échappent au dispositif d'échange de données toutes les administrations qui se trouvent dans l'« impossibilité technique » d'échanger. Il n'est donc pas utile d'exempter les collectivités de moins de 10 000 habitants

restriction est assez peu compréhensible dans la mesure où ce dispositif d'échange de données existe depuis 2015, sans qu'il ait été révélé de difficultés pour les communes de moins de 10 000 habitants.

sous couvert de ne pas charger les communes de tâches supplémentaires, de pénaliser les habitants des territoires ruraux, qui sont souvent les plus éloignés de l'administration

» est strictement limité à l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires.

des échanges d'informations ou de données. C'est en ce sens que j'avais déposé un amendement en commission, à la suite de nombreux retours de maires, notamment de mon département du Bas-Rhin.

tend à préciser que le décret en Conseil d'État prévu à l'article 50 encadrera les cas dans lesquels les communes pourraient avoir à connaître d'informations relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

est à M. Éric Kerrouche. À l'article 50, le Gouvernement propose de mettre en place un échange d'informations ou de données entre administrations, afin d'informer les personnes sur leurs droits au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévu par la loi.

et les traitements mis en oeuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d'une fraude. » Je pense qu'il s'agit d'une erreur de plume et que les

de l'analyse du Conseil d'État. Dès lors que les échanges de données concernent par hypothèse des usagers n'ayant pas présenté de demande ou de déclaration à l'administration, donc n'ayant pas consenti à l'utilisation de leurs données,

: La parole est à M. Patrick Chaize. La notion de données d'intérêt général, instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, vise à permettre aux autorités publiques d'obtenir la communication ou de publier certaines données détenues par des personnes de droit privé dès lors qu'elles sont utiles à l'exercice de leurs compétences ou à l'information des citoyens. Sans donner de définition générale de ces données, la loi renvoie à certaines catégories spécifiques et, en particulier, aux données liées aux contrats de concession de service public, ainsi qu'aux données essentielles des conventions de subvention conclues par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial. Toutefois, en pratique, d'autres données détenues par des personnes morales de droit privé peuvent être très utiles à l'élaboration, à la mise en oeuvre ou à l'évaluation d'une politique publique locale alors même que lesdites personnes morales de droit privé ne sont pas liées contractuellement aux collectivités et groupements de collectivités concernés. Il convient donc que ces collectivités et groupements de collectivités bénéficient d'une certaine souplesse en définissant au cas par cas, et selon une délibération motivée tenant compte des politiques publiques mises en oeuvre sur leur territoire, la liste des données et des bases de données privées qui peuvent présenter un caractère d'intérêt général. Il est donc proposé d'habiliter les collectivités territoriales et leurs groupements à délibérer pour définir, chacun en ce qui le concerne, la liste des données et des bases de données privées d'intérêt général au regard des politiques publiques locales qu'ils mettent en oeuvre, et selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

une liste de données privées d'intérêt général qui seraient nécessaires à l'exercice de leurs compétences et qu'elles seraient en droit de demander à toute personne morale

loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, vise en effet les données privées dont la publication peut se justifier en raison de leur intérêt pour améliorer les politiques publiques. Toutefois, ne sont concernées que les données privées issues des contrats de concession ou de délégation de service public, les données essentielles des contrats de subventions et certaines données de personnes morales de droit privé, à des fins exclusives d'établissement de statistiques. Il est donc très délicat d'élargir le dispositif en permettant aux collectivités de solliciter directement la communication de données privées. La mesure proposée risquerait d'être inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété, aux libertés économiques et aux libertés individuelles.

telle disposition a d'ailleurs été adoptée à deux reprises par le Sénat. Elle a ainsi été votée par la Haute Assemblée dans le cadre du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, puis supprimée par l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a une nouvelle fois adoptée le 16 janvier 2020 dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale. Ce texte, initié par Sylvie Vermeillet et Hervé Maurey, n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale. Le droit à régularisation d'une erreur a été reconnu pour tout usager de l'administration, entreprise ou particulier, qui méconnaîtrait involontairement et pour la première fois une règle applicable à sa situation sans faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou être privé d'une prestation due. Il ne s'applique toutefois pas aux collectivités locales. Pourtant, ce serait pleinement justifié. Le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter. La situation est aggravée par la baisse de leurs ressources sous l'effet de la diminution des dotations, qui les a contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d'autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l'État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d'appui juridique des collectivités locales. Or les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment les plus petites. Cet amendement vise à étendre le droit à l'erreur prévu pour les entreprises et les particuliers aux collectivités locales et à instituer un droit à régularisation spécifique

les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient déjà, en tant qu'employeurs, des mesures protectrices du code de la sécurité sociale

En outre, l'amendement est d'ores et déjà satisfait par le régime juridique actuel des demandes de subventions au titre des dotations de l'État, qui est favorable aux collectivités territoriales : si l'incomplétude du dossier n'est pas signalée aux demandeurs,

s'appliquerait même en cas de méconnaissance des règles applicables et d'erreurs matérielles présentant un caractère répété. À l'inverse, le droit à l'erreur dont peuvent bénéficier les particuliers

la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) visés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques (SDUSN), qui permet de coordonner les différentes offres de services numériques sur un territoire et d'en faciliter leur développement. Un certain nombre de ces services portent sur des données de référence au sens de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. La SDUSN doit donc pouvoir être utilisée par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leur permettre de contribuer au service public des données de référence, comme le prévoit la loi. C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser le contenu de la SDUSN, de manière à faire de cet outil de planification locale un moyen de mise en oeuvre dans les territoires du service public des données de référence. Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des attaques par rançongiciels visant en particulier les activités de service public gérées par les collectivités territoriales et leurs groupements, il est important d'intégrer dans la stratégie des services numériques menée au niveau local les actions visant à renforcer la cybersécurité desdits services.

que la gestion des données et la cybersécurité deviennent progressivement un enjeu incontournable ; vous avez rappelé les attaques récentes. Pour autant, il me paraissait prématuré d'imposer aux collectivités territoriales d'intégrer ces enjeux dans leurs schémas de manière obligatoire et de devoir les réviser. Une telle obligation se serait appliquée un peu difficilement. Vous avez bien voulu transformer

Depuis la réforme de 2016, la fin du principe de territorialisation des demandes a encore ajouté de l'incompréhension chez les habitants. Désormais, ils doivent se rendre dans une commune équipée d'une station de recueil non seulement pour effectuer leur demande, mais aussi pour retirer leur nouveau titre d'identité. en zone rurale, peu de communes disposent d'un tel équipement. Les personnes devant accomplir cette démarche doivent donc se rendre dans une autre mairie, souvent éloignée de leur domicile. La crise sanitaire a plus que jamais démontré que c'est vers les maires et leurs équipes que les administrés se tournent

Cette tâche constitue un service de proximité essentiel et fait partie des missions permettant aux communes d'établir et de maintenir un lien avec la population, qui est très utile au quotidien. beaucoup d'élus souhaitent pouvoir de nouveau assurer ce service de proximité. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet article additionnel permettant aux communes qui souhaitent reprendre cette compétence d'être mises en relation avec les communes qui disposent d'appareils

la mise en place de hubs territoriaux sur la base d'appels à projets qui ont obtenu des réponses très disparates à travers le pays.

Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.

confrontés à un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui, face à la dématérialisation croissante des procédures administratives et à l'irruption du numérique dans leur vie quotidienne, se trouvent désarçonnés et en difficulté.

pour le faire, mais il nous semble important et urgent de donner une valeur législative à ces schémas et d'encourager l'ensemble des départements à se saisir de cette question et à s'engager dans cette voie. Les cinq amendements suivants sont

à l'échelle des départements soit une solution. Il est préférable de faire confiance aux collectivités, plutôt que de les soumettre à des carcans administratifs qui s'accumulent au fil des ans.